Dès l'année 2018, et jusqu'en 2021, la droite propose que le taux du versement transport augmente de 0,21 point par an, pour passer de 2,12 % en 2017 à 2,95 % en 2021. Au premier abord, cet article peut paraître répondre au rétablissement d'une certaine équité entre les départements en matière de versement transport. Mais, en réalité, la logique de cet article est mortifère : elle revient à aggraver encore le déséquilibre emploi-habitat entre l'est et l'ouest franciliens, en portant un coup au développement économique de ces deux départements populaires. Il faudrait trouver, au contraire, des mesures incitatives permettant de faire reculer ces inégalités criantes, tout en mobilisant de nouvelles ressources pour le financement des transports publics en Île-de-France. Dans cet esprit, nous proposons, et ce depuis de nombreuses années, d'augmenter les taux du versement transport dans les Hauts-de-Seine et dans certains quartiers de Paris, bien dotés en réseaux de transport et abritant de nombreuses entreprises. Plus précisément, nous proposons de porter ce taux à 3,5 % dans les Hauts-de-Seine et à Paris, ... Ben tiens ! ... à l'exception des communes et arrondissements les plus pauvres. N'est-ce pas plus juste territorialement et économiquement ? Pour rappel, Paris et les Hauts-de-Seine totalisent plus de 55 % de l'offre de mètres carrés de bureaux en Île-de-France. La tendance ne fait d'ailleurs que s'accentuer, comme le confirment les chiffres de l'Observatoire régional de l'immobilier d'entreprise, avec des emplois qui ne se sont jamais autant polarisés que dans ces zones. Or tout est lié. Chacun sait que l'engorgement des transports en commun résulte de l'aménagement du territoire, avec une concentration des bureaux à l'ouest et de l'habitat à l'est. Autre élément qui plaide pour notre amendement, les recettes récoltées s'élèveraient à 350 millions d'euros par an, ce qui n'est pas négligeable. Elles permettraient, par exemple, à Mme Pécresse, présidente du conseil régional d'Île-de-France et d'Île-de-France Mobilités, de disposer de marges financières suffisantes pour ne pas augmenter pour la troisième fois consécutive les tarifs

profondeur. Les élus locaux doivent bénéficier d'un statut leur permettant d'assumer leurs responsabilités pleinement et dignement. Cet amendement ne vise pas, néanmoins, à entrer dans ce débat aujourd'hui ; il tend seulement à corriger de manière concise et efficace une anomalie législative. chers collègues, les présidents d'exécutifs locaux, les conseillers régionaux et conseillers départementaux ont vu leurs fonctions profondément modifiées par les différentes lois de réforme territoriale. La loi NOTRe a confié au président de région des compétences stratégiques essentielles, qu'il s'agisse du développement économique, de la gestion des programmes européens, de la formation professionnelle ou encore de l'aménagement du territoire ou des transports. Quant au président du conseil départemental, il est responsable des solidarités et de la cohésion territoriale, missions de haute importance, et dont nos territoires ont plus que jamais besoin. Nous devons donc reconnaître ces très lourdes responsabilités qui pèsent sur les présidents des exécutifs locaux. Qui peut prétendre que l'exercice d'une telle fonction n'est pas comparable à un poste à forte responsabilité au sein de la haute fonction publique ? Le montant maximal que peut toucher un président de région est aujourd'hui bien inférieur à celui de ses propres collaborateurs. Je n'ai pas besoin de vous faire l'inventaire des rémunérations de la haute fonction publique, qui, avec les primes et l'ancienneté, atteignent des montants bien plus importants. Cet amendement a pour objet de corriger cette anomalie et d'accorder une véritable reconnaissance aux responsabilités et au travail exigeant des chefs d'exécutifs locaux.

Il s'agit tout simplement, et bien naturellement, de reconnaître le travail et l'engagement des élus locaux.

les logements qui font l'objet d'une opération de rénovation urbaine. Vous proposez, par cet amendement, de sortir du champ de l'exonération les bâtiments qui ont déjà profité, lors d'un programme précédent, d'une exonération plus longue. La mécanique peut s'entendre. C'est pourquoi le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

tour ! Au bout du compte, en effet, ce sont les communes qui paient l'addition. Cela fait longtemps que j'appelle de mes voeux une remise à plat de tout ce système. Il peut y avoir de bonnes raisons d'exonérer les bailleurs sociaux, ne serait-ce que pour les aider,

d'euros, y compris le fonds d'aide à la rénovation thermique pour un montant de 80 millions d'euros. Ils se répartissent de la manière suivante : 512,1 millions d'euros aux propriétaires pour le financement de leurs travaux ; 6,2 millions d'euros à l'humanisation des structures d'hébergement ; 52,2 millions d'euros à l'ingénierie ; 11,5 millions d'euros aux opérations de résorption de l'habitat insalubre. Ces aides ont permis d'engager un volume de travaux éligibles de 1,26 milliard d'euros, soit l'équivalent de 21 000 emplois créés ou préservés. Au total, 69 769 logements sont rénovés grâce à ces aides : 56 615 logements dans le cadre d'aides directes aux propriétaires ; plus de 13 000 logements au travers de 361 syndicats de copropriétaires ; 137 logements dans le cadre d'aides dédiées aux communes, c'est-à-dire

ou l'extension de bâtiments existants. Cette exonération est déjà large, puisqu'elle peut concerner les ventes en l'état futur d'achèvement dans les constructions nouvelles, mais aussi les opérations de reconstruction ou les additions de constructions.

aux immobilisations industrielles en matière de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises. Faute de définition légale de la notion d'immobilisation industrielle, l'administration fiscale en fait une interprétation extensive l'autorisant à soumettre à ce régime tout établissement « où le rôle de l'outillage et de la force motrice est prépondérant ». Nombre d'entreprises artisanales voient malheureusement leurs locaux requalifiés en locaux industriels, avec une augmentation de leur cotisation foncière pouvant aller jusqu'à 300 %.

pour présenter l'amendement n° II-501 rectifié. Cet amendement vise à instituer une « taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés » qui serait le fruit de la fusion de deux taxes, à savoir la taxe sur les logements vacants et la majoration de taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Dans un contexte de disparition programmée de la taxe d'habitation, cette nouvelle taxe permettrait de sécuriser juridiquement les politiques de lutte contre la captation d'une partie des logements par des résidences secondaires ou des locations meublées de courte durée, captation croissante dans les communes situées en zone tendue. En effet, chaque année, des milliers de logements du parc des résidences principales disparaissent, entravant ainsi l'accès au logement pour la population résidante, déséquilibrant la vie et l'économie de quartiers entiers, et limitant l'efficacité des outils classiques de la politique du logement. Grâce à cette taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés, les communes des zones tendues seront dotées d'un levier fiscal réellement efficace, permettant d'adapter le niveau de taxation aux problématiques locales. Cet amendement ne remet en cause ni la taxe prévue à l'article 232 du code général des impôts ni le système de plafonnement actuel du taux de la taxe d'habitation, qui concerne ces logements et qui garantit une juste proportionnalité de l'imposition.

Dans la seule agglomération parisienne, plus de 300 000 logements soit sont vacants, soit sont des résidences secondaires occupées, pour la plupart, moins d'une semaine à l'année. Il est indispensable de mieux mobiliser cette offre vide ou très peu occupée, ce qui permettrait d'offrir très rapidement des centaines de milliers de logements supplémentaires

dirigées par des élus de toutes sensibilités politiques. Mais du fait de la coexistence d'une taxe sur les logements vacants et d'une autre sur les résidences secondaires, il est parfois plus profitable de laisser son logement vacant. Afin de doter les communes des zones tendues d'un levier fiscal réellement efficace, permettant d'adapter le niveau de taxation aux problématiques locales, cet amendement tend à fusionner la taxe d'habitation sur les résidences secondaires applicable aux zones tendues et la taxe d'habitation sur les logements vacants. La taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés en zone tendue ainsi créée sera un outil clair, lisible, efficace, simple et immédiatement opérationnel pour mobiliser des centaines de milliers de logements. Elle permettra à autant de ménages d'accéder plus facilement à un logement, et contribuera à exercer une pression à la baisse sur les niveaux de loyer.

puisque votre proposition se traduirait par des superpositions d'impositions différentes, là où une seule taxe est actuellement applicable. Pour les résidences secondaires situées dans les agglomérations de plus de 50 000 habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, la nouvelle taxe s'ajouterait à la Pour les logements vacants situés dans ces mêmes zones, elle s'ajouterait à la taxe sur les logements vacants prévue à l'article 232 du code général des impôts. Enfin, cette mesure aurait pour conséquence d'augmenter très fortement

l'assimilation des centres de pressurage et des petites installations de vinification à des établissements industriels entraîne l'application de la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code du code général des impôts lorsque les locaux sont inscrits à l'actif d'un bilan réel. L'assiette ainsi déterminée ne bénéficie pas du coefficient de neutralisation mis en place dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels. Les bases d'imposition des locaux entrant dans le champ de la méthode comptable sont donc considérablement supérieures à celles qui résultent de l'application des valeurs locatives révisées, toutes choses égales par ailleurs. Afin d'éviter l'inégalité de traitement pour les locaux utilisés par de petites entreprises, il est proposé d'exclure du champ d'application de la méthode dite « comptable » les locaux dont la valeur brute est inférieure à 2 millions d'euros.

Ces locaux sont assimilés par l'administration fiscale à des établissements industriels. L'imposition, qui repose, dans ce cas, sur la valeur brute des bâtiments et non sur l'importance de l'activité qui y est exercée, est particulièrement lourde et pénalisante pour les bâtiments abritant des activités qui ne s'exercent que quelques semaines par an,

d'étendre à ces locaux les dispositions applicables aux locaux servant à l'hébergement des salariés saisonniers, par le calcul de la base d'imposition au prorata du temps d'utilisation des locaux à la réalisation de l'activité saisonnière. Bien entendu, cette réduction de la base d'imposition

parce que tout l'équilibre d'un secteur économique est en jeu au travers de ces simples dispositions.

à l'exonération de la taxe sur les surfaces commerciales applicable aux établissements ouverts avant le 1 janvier 1960. Cette disposition est désormais, surtout pour les établissements repris depuis cette date, impropre à tenir compte des situations de concurrence commerciale comme de la réalité de l'évolution urbaine et des fréquentations touristiques. Je donnerai un seul exemple : nombre de commerces de centre-ville historiquement installés, ouverts avant 1960, ne paient aujourd'hui pas la TASCOM. C'est notamment le cas, à Bordeaux, d'une grande enseigne vestimentaire qui a tout à fait les moyens de payer cette taxe. La situation actuelle est particulièrement injuste et elle est de nature à fausser la concurrence.

Ces dispositions ne permettent pas d'intégrer dans l'assiette de la TASCOM les points de distribution de marchandises de type, car ceux-ci ne sont pas nécessairement considérés comme appartenant à un ensemble commercial. Il est grand temps d'y remédier, et c'est précisément ce à quoi tend cet amendement. Nous en avons déjà largement parlé

concernant la TASCOM. Il s'agit ici d'adapter le champ d'application de la TASCOM pour éviter les pratiques d'optimisation fiscale, telles que la signature de contrats de location-gérance, pratiques non visées par la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés. Une disposition de la loi précitée intègre, dans le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales, les installations de vente au détail de carburant des établissements soumis à la taxe, lorsque soit l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants, soit l'établissement contrôle directement ou indirectement une installation de distribution au détail de carburants, soit l'établissement et une installation de distribution au détail de carburants sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne. L'intention du législateur, au-delà de ces précisions, consistait à bien intégrer dans l'assiette de calcul de la taxe cette activité commerciale spécifique. Or il s'avère que certains contribuables- c'est le cas dans la communauté urbaine de Bordeaux -recherchent des possibilités d'optimisation fiscale en établissant des formes de gestion non visées par l'article 3, alinéas 9 et 11, de la loi précitée, tels des contrats de location-gérance, qui ne sont pas assimilables à du contrôle direct

? Vous me pardonnerez, madame Delattre, mais le Gouvernement n'est pas favorable à mesure que vous proposez. Vous voulez majorer le taux de la TASCOM applicable aux magasins de vente au détail lorsque, sur le même site, il existe une installation de vente au détail de carburant exploité par un tiers.

Votre intention est de prendre en compte l'activité de vente de carburant pour majorer le tarif ou l'assiette de la taxe, lorsque le magasin de vente au détail redevable de la TASCOM exerce un certain contrôle sur cette activité,

pour déclarer le dossier complet- deux mois pour notifier les éventuelles pièces manquantes et deux mois pour compléter le dossier. Ainsi, très concrètement, pour nos collègues qui ne comprendraient pas grand-chose à ce que je dis, cela veut dire que l'amendement permet d'éviter que des communes

l'avis du Gouvernement ? Le Gouvernement n'a pas tout à fait la même position que la commission sur le sujet. Ah ! ... D'abord, je veux rappeler que les pièces constitutives du dossier de demande de classement sont détaillées dans la circulaire du 3 décembre 2009 relative aux communes touristiques et aux stations classées supposer que, depuis 2009, connaissance a été prise de cette liste de pièces. Le dépôt d'un dossier complet est plus qu'une formalité administrative, il traduit la maturité de la démarche engagée par la commune pour obtenir, dans le cas d'espèce, son classement ; et, si le dossier est effectivement complet au moment du dépôt, les services du préfet peuvent délivrer une attestation dès réception. Ce n'est qu'en raison de l'absence, dans le dossier de demande de classement, de certaines pièces indispensables- par exemple, l'arrêté de classement de l'office du tourisme, la capacité d'hébergement suffisante ou encore l'absence de signalement, par l'agence régionale de santé, -que le certificat de complétude ne peut être délivré. Dans la plupart des cas, lorsque le dossier a été travaillé en amont par la collectivité, la délivrance du certificat est extrêmement rapide. En outre, amender l'article 45 dans le sens que vous proposez créerait un appel d'air vis-à-vis de toutes les communes qui n'ont pas anticipé les délais de renouvellement de leur classement, pourtant connus depuis l'entrée en vigueur de la réforme, le 3 mars 2009. Cela pourrait donc dénaturer le principe même du classement en station de tourisme comme label d'excellence touristique.

alors que les biens loués peuvent être, dans les faits, d'une catégorie bien supérieure. Afin de rétablir une équité fiscale entre les hébergeurs classés est donc proposé d'offrir la possibilité aux collectivités qui le souhaitent d'appliquer à ces meublés non classés une taxation proportionnelle au prix de la chambre, dans la limite de 3 %. Ainsi la taxe de séjour acquittée serait bien, pour ces établissements non classés, proportionnelle à la qualité

On peut déjà convenir d'une chose : le barème de la taxe de séjour est imparfait. D'ailleurs, nous serons amenés à l'étudier à la fin de la semaine, vendredi ou samedi, puisque,

Pourquoi ? Parce que la taxe de séjour unique peut avoir des effets négatifs sur la fréquentation touristique de certaines communes, notamment rurales, qui n'ont pas nécessairement les mêmes outils, les mêmes infrastructures, ni les mêmes capacités que les communes touristiques

au nom de la délégation aux entreprises. La loi de finances pour 2016 a instauré l'obligation d'utiliser, à compter du 1 janvier 2018, un logiciel de comptabilité ou de gestion, un système de caisse conforme à des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage. Le présent article limite cette obligation aux seuls logiciels et systèmes de caisse, qui sont les principaux vecteurs des fraudes constatées à la TVA. Cet amendement amendement a un double objectif. D'une part, il vise à reporter la mise en application de la mesure d'un an, au 1 janvier 2019, afin de laisser le temps aux entreprises de s'adapter au vu de la situation actuelle, une grande majorité d'entreprises ne seront pas en capacité d'être prêtes au 1 janvier 2018. D'autre part, il tend à imposer aux fournisseurs d'équipement, fabricants ou éditeurs de logiciel, qui sont responsables de la certification, d'émettre l'attestation de conformité au moment de l'installation, afin d'éviter la complexité administrative que représente pour les petites entreprises le fait de courir après l'attestation.

l'attestation. Il est donc essentiel que la responsabilité de la délivrance de l'attestation soit assumée par les fournisseurs de matériel, et que les commerçants de proximité ne subissent ni l'insécurité juridique

Il est donc proposé que les vendeurs présents sur ces plateformes puissent présenter, en lieu et place du certificat portant sur le système de gestion des encaissements, le document récapitulant le montant des transactions.

l'avis du Gouvernement ? La fraude à la TVA par la dissimulation de recettes a été effectivement facilitée par la commercialisation de logiciels ou systèmes de caisse frauduleux, qui permettent d'effacer des recettes et de reconstituer les tickets de caisse sans que cette manipulation soit décelable. Les certificats demandés dans le cadre du présent article s'appliquent au système de gestion des règlements encaissés par une entreprise pour son activité propre, qu'il s'agisse de vente ou de prestation de services auprès de clients particuliers et quelle que soit la modalité de vente, physique ou en ligne. Les sociétés du e-commerce relèvent donc du champ d'application du dispositif. Il n'y a pas de raison d'établir un régime de faveur à leur égard. En effet, le Gouvernement rappelle que les modalités de l'encaissement des paiements ne sont pas nécessairement plus sécurisées dans ce secteur que dans d'autres. Par exemple, la perception de loyers des cartes prépayées n'est pas vraiment un gage de transparence. Par ailleurs, la simplification proposée ne paraît pas appropriée, car le document récapitulant le montant brut des transactions effectuées une plateforme n'a pas le même objet et n'offre pas les mêmes garanties que la sécurisation des systèmes de caisse. Le document visé est un simple récapitulatif annuel, qui ne garantit ni la traçabilité des encaissements, ni leur inaltérabilité, ni leur archivage. Il ne répond donc pas aux conditions fixées par la loi. Par ailleurs, les dispositions n'allégeraient pas les obligations incombant aux petits commerçants qui ont à la fois une boutique physique et une boutique en ligne, qui devraient en tout état de cause faire certifier ou attester de la sécurité de leur logiciel ou système de caisse. Dans ces conditions, le Gouvernement sollicite le retrait de l'amendement.

en 2022. Ce projet permet aux entreprises de bénéficier d'un taux d'IS à 28 % dès 2018 sur les cinq cents premiers milliers d'euros de bénéfices et d'améliorer ainsi leur santé financière et leur compétitivité. Toutefois, ce projet d'abaissement de la taxation des entreprises ne concerne que l'impôt sur les sociétés et délaisse ainsi plus de 50 % des entreprises, qui sont imposées à l'impôt sur le revenu et qui attendent elles aussi des gains de compétitivité et de rentabilité par un allégement de la fiscalité pesant sur elles. C'est pourquoi le présent amendement vise à proposer une mesure de baisse d'impôt en faveur de ces entreprises, à travers la suppression de la majoration de 25 % des revenus des entreprises

l'avis du Gouvernement ? Le Gouvernement partageait les interrogations de M. le rapporteur général sur le caractère législatif ou réglementaire de certaines dispositions. D'ailleurs, il avait fait état de ses doutes lors de l'adoption de l'article à l'Assemblée nationale. Depuis, un travail de concertation

à éviter de mettre en place une sorte de tactique fiscale qui mettrait en difficulté soit les enseignes de proximité, soit les usagers cédant des biens d'occasion, dont je rappelle qu'ils sont exonérés de TVA à hauteur de 3 000 euros par an.

qui m'amènent à dire que la France est impliquée de manière très active dans le lancement et la conduite du projet de lutte contre l'optimisation fiscale de l'OCDE, le plan d'action BEPS. Par ailleurs, elle a signé le 7 juin 2017, avec plus de 70 la convention multilatérale qui traduira les conclusions de ces travaux dans les conventions fiscales bilatérales de la France et des autres signataires. L'une des dispositions de cet accord vise notamment à lutter contre les montages de commissionnaires visés par ces amendements. Cet objectif sera donc traduit dans les conventions fiscales bilatérales de la France à la suite de la signature de l'accord.

qui offrent à l'administration fiscale des moyens équivalents, sinon plus efficaces. On peut citer l'abus de droit, prévu à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, qui permet de remettre en cause les montages dépourvus de substance économique et qui est assorti d'une pénalité de 80 %. De plus, la loi prévoit un renversement de la charge de la preuve pour la déduction de la totalité des dépenses réalisées en direction d'un territoire à faible fiscalité, tel que défini à l'article 238 A du code général des impôts. Enfin, nous disposons également d'une procédure qui permet d'imposer les bénéfices d'un établissement stable non déclaré sur notre territoire. Nous considérons qu'il ne faut pas doublonner ces outils ni, surtout, remettre en cause leur utilisation et la traduction de l'accord du 7 juin 2017. Enfin, concernant la fiscalité du numérique et des activités conduites sur internet, nous considérons que les niveaux européen et mondial sont plus adaptés. C'est à ces échelons qu'agit le Gouvernement. Gouvernement. La France a récemment obtenu une accélération décisive, à l'occasion du conseil ECOFIN informel de Tallinn, qui s'est tenu les 15 et 16 septembre, puis le 5 décembre dernier, avec des conclusions sur une approche commune des ministres

fin de 2015 a probablement eu quelque effet sur la politique du gouvernement en 2016 et en 2017, notamment sur les différents éléments que vous avez rappelés. Pour autant, nous sommes bien obligés de constater qu'une décision du tribunal administratif dit, en gros, que l'État

Ces contributions prennent le plus souvent la forme de rémunérations de prestations de services excédant la valeur réelle de ces dernières, voire relatives à des prestations fictives. Il en est de même des redevances. Ces centrales sont établies dans des pays à fiscalité réduite, de sorte qu'une partie significative d'assiette fiscale se trouve délocalisée, au détriment des finances publiques, sans justification. Le présent amendement vise notamment à réintégrer le montant de ces prestations ou redevances dans les bénéfices ou revenus imposables des distributeurs, dès lors que les produits livrés par les industriels, et au titre desquels sont rémunérées ces prestations, ou sur la base desquels sont déterminées les redevances, sont mis sur le marché dans une surface de vente implantée en France. Contrairement à ce qui a pu être dit lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2017, cet amendement se distingue, à plusieurs égards, des dispositions existantes.

Aucun seuil de détention minimal n'est fixé s'agissant des relations capitalistiques. Le dispositif de cet amendement vise, plus précisément, les sociétés françaises exploitant des magasins ou des établissements de vente en France liées à des centrales à l'étranger. il vise les sociétés françaises parties à un ou à des accords d'achats groupés avec des entreprises ou entités juridiques établies à l'étranger. Enfin, aucune limitation aux entités établies dans un pays à régime fiscal privilégié n'est prévue. De plus, les dispositions de cet amendement visent des revenus spécifiques, alors que l'article 209 B

qui regrette de ne pouvoir être présent pour le défendre tant l'enjeu est important. Il s'agit d'un amendement anti-optimisation fiscale des réseaux de la grande distribution. Le sujet est complexe, mais l'objet de l'amendement répond avec précision aux arguments avancés par Bercy. À l'heure actuelle, les distributeurs À l'heure actuelle, les distributeurs exigent que des contributions soient versées à leurs centrales situées en Europe. Ces contributions prennent la forme de rémunérations de prestations de services excédant la valeur réelle de ces voire relatives à des prestations fictives. Il en est de même des redevances, dont on ne sait pas très bien à quoi elles correspondent. Les centrales captant ces revenus sont établies dans des pays à fiscalité réduite- essentiellement au Luxembourg, en Suisse et en Belgique de sorte qu'une partie significative d'assiette fiscale se trouve délocalisée, au détriment des finances publiques, sans que cette délocalisation soit justifiée par une activité effective. Le présent amendement vise donc à réintégrer le montant de ces prestations ou redevances dans les bénéfices ou revenus imposables des distributeurs, dès lors que les produits livrés par les industriels sont mis sur le marché dans une surface de vente située en France. Par ailleurs, il semblerait qu'une directive européenne couvrant les cas visés par les dispositions de cet amendement soit prochainement transposée. Merci,

l'article 209 B du code général des impôts impose les bénéfices d'entités détenues de façon directe ou indirecte depuis la France et établies dans un État étranger, où elles présentent une imposition réduite, voire nulle. Ce dispositif anti-abus permet de couvrir les situations de délocalisations fictives ou abusives. En deuxième lieu, dans une logique de prix de transfert, l'article 57 du code général des impôts exige que les conditions convenues dans le cadre de leurs relations financières ou commerciales par des parties dépendantes soient celles auxquelles on pourrait s'attendre si les parties n'avaient aucun lien de dépendance. La notion de dépendance peut être juridique ou de fait ; elle n'est pas limitée à des relations capitalistiques et peut résulter d'un contrat ou des conditions dans lesquelles s'établissent les relations entre deux entreprises. Ainsi ce dispositif permet-il d'appréhender une situation éventuelle de transferts de bénéfices similaire à celles visées dans le cas des centrales d'achat. Sur le fondement de l'acte anormal de gestion, les services de contrôle peuvent remettre en cause la déduction en charges, par une entreprise, d'une commission payée à une autre si cette opération ne répond pas à l'intérêt de l'exploitation. En troisième lieu, comme vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur général, ces mêmes services peuvent recourir à la procédure de l'abus de droit fiscal, prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.

Monsieur le secrétaire d'État, mercredi 6 décembre, dans ce même hémicycle, à l'occasion de l'examen de la mission « Crédits non répartis », vous êtes revenu sur la prime de compensation de la hausse de la CSG pour les agents publics publics : « Depuis le 30 novembre dernier, le Conseil national d'évaluation des normes a été saisi d'un décret permettant l'abaissement de la cotisation employeur maladie de 11,5 % à 9,9 %. Ainsi, d'un point de vue macroéconomique, l'intégralité des coûts liés à la hausse de la CSG

Mais au niveau microéconomique, pouvez-vous nous garantir la neutralité de l'augmentation de la CSG pour les employeurs, comme vous souhaitez la garantir pour l'ensemble des fonctionnaires touchés par cette mesure ? » Le mot « microéconomique » est ici essentiel. Je vais vous donner quelques exemples. Pour un agent titulaire effectuant plus de 28 heures par semaine et payé à l'indice majoré 320, la perte pour la collectivité est de 9,23 euros par mois pour un agent titulaire effectuant plus de 28 heures par semaine, payé à l'indice majoré 360, la collectivité gagne 10,17 euros par mois. Pour un agent contractuel ou un agent titulaire à temps non complet effectuant moins de 28 heures par semaine, payé à l'indice majoré 320, la collectivité perd 25,04 euros par mois

124 paragraphe II, le dispositif de la TVA à taux réduit à certaines opérations de travaux aux établissements hébergeant des enfants handicapés. Par ailleurs, la loi dite DALO a fondé le bénéfice de la TVA à taux réduit pour les opérations de travaux conduits

Le champ des établissements accueillant des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans au titre de l'aide sociale à l'enfance n'était quant à lui pas concerné par cette mesure de soutien à l'investissement et aux opérations de rénovation et mises en conformité. Le présent amendement vise donc à harmoniser les taux de TVA applicables dans l'ensemble des établissements sociaux et médico-sociaux destinés à l'hébergement des enfants. L'amendement

de préciser que les deux tiers des salariés ne restent pas sans aucune rémunération pendant ces trois jours de carence, puisque, dans de nombreuses entreprises, la convention collective prévoit que c'est l'entreprise qui prend à sa charge une partie ou la totalité de cette période de carence. Je rappelle que, en 2012, le gouvernement de M. Sarkozy avait mis en place le jour de carence dans la fonction publique. Il a été supprimé en 2014, son impact sur les dépenses de l'assurance maladie ayant été considéré comme négligeable. Une note récente de l'INSEE note récente de l'INSEE montre que, entre 2012 et 2014, le jour de carence n'a pas significativement modifié la proportion d'agents de la fonction publique de l'État absents pour raison de santé. Cette mesure s'est même avérée contre-productive, si les absences pour raison de santé de deux jours ont diminué, les absences d'une semaine à trois mois ont augmenté durant la même période. Enfin, l'INSEE précise que le nombre d'absences courtes a davantage diminué dans certaines les jeunes et les employés travaillant peu de jours par semaine, qui ont pu prendre sur leurs jours chômés pour se soigner. En conclusion, je tiens à dire que le rétablissement d'un système inefficace et injuste est un mauvais coup supplémentaire qui s'abat sur la tête des fonctionnaires, lesquels sont bien les sacrifiés

aucune action de prévention au cours des douze derniers mois : manque de moyens ou manque de compétences en interne, les raisons sont multiples. La lutte contre l'absentéisme n'a de sens que si le lien est fait entre absences pour raisons de santé et exposition à des risques professionnels ou psychosociaux. C'est une approche globale du sujet qu'il faut envisager et non une mesure stigmatisante

Le scrutin est ouvert.

Je leur suggère de soutenir la natalité en donnant aux femmes enceintes les conditions sanitaires appropriées à leur état. Je ne crois pas qu'on puisse apporter une réponse à cette question par les congés de grossesse pathologique. Il s'agit au contraire d'éviter que les femmes

relèvent de conventions collectives qui ne prévoient pas de jours de carence, grâce à la mensualisation. On parle donc d'aligner le régime des fonctionnaires sur le régime d'un tiers des salariés du privé,

Dans ce cas, il ne faut pas pousser les femmes à recourir à des congés maladie ! Pas un seul médecin ne refuserait à une femme enceinte qui se dit

cet amendement rejoignent celles qui ont été votées tout à l'heure pour ce qui concerne les GAFA. Afin d'inclure dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés en France par les entreprises numériques, dont l'activité est par nature évanescente, il est proposé d'introduire

les conventions fiscales internationales, le Sénat et l'Assemblée nationale n'interviennent qu'à la fumée des cierges, une fois qu'elles ont été signées. Et elles ne peuvent pas être amendées ! Nous avons eu ici plusieurs débats très intéressants sur l'efficacité des conventions fiscales internationales. Toutefois, le Parlement n'a absolument aucune

dans le débat ... -, mais oublie les poids lourds de l'optimisation fiscale, à commencer par ceux qui se trouvent au sein même de l'Union européenne.

Pourquoi donc un tel aveuglement ? L'évasion et la fraude fiscales menacent pourtant directement les économies européennes et mondiales. Le manque à gagner, en Europe, est évalué à 1 000 milliards, dont 70 à 80 milliards pour la France. C'est l'équivalent de notre déficit public ! Il est urgent de se donner les moyens de punir ceux qui, en cherchant à s'affranchir de l'impôt, refusent de payer le prix de la civilisation et de la solidarité. Nous ne pouvons donc, en France, que nous émanciper des orientations de la Commission européenne, ... Il faut conclure, cher

et inscrire une obligation de débat dans la loi serait trop rigide. Concernant la publication du rapport annuel sur le réseau conventionnel de la France en matière d'échange de renseignements, puisqu'il s'agit de cela, en effet, pour des raisons visiblement liées à l'agenda, ces rapports n'ont pu être présentés ni en 2014, ni en 2015, ni en 2016. Aussi, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous propose de vous transmettre un document à jour des données de 2017 au cours des prochains mois, en complément des réponses que nous avons apportées au récent questionnaire de la commission des finances.

États-Unis, au Canada, en Irlande. En cas de défaut de déclaration préalable, le schéma d'optimisation fiscale ne serait pas opposable à l'administration fiscale.

un marronnier ! Personne ne l'ignore ici : les affaires de fraude, qui sont susceptibles de faire l'objet de poursuites pénales, sont soumises depuis quarante ans à un régime particulier, celui de leur examen par la Commission des infractions fiscales, autorité administrative indépendante traitant environ un millier de dossiers sensibles par an.

de tenter de mettre fin à des confusions qui peuvent parfois être entretenues. Il y a le verrou de Bercy, tel qu'on le dénomme communément ; il y a un certain nombre de procédures, rares,

plaide coupable d'une infraction, notamment de blanchiment. Une telle convention de règlement est intervenue récemment entre le Parquet national financier et la société HSBC dans le cadre d'une affaire de blanchiment. Il faut préciser que, dans ce dernier cas- il s'agissait de

Lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2016, les députés avaient proposé d'introduire, à compter du 1 janvier 2017, l'obligation pour les plateformes numériques collaboratives de communiquer à l'administration fiscale les revenus perçus par leurs utilisateurs. En améliorant l'information de l'administration fiscale, l'objectif était tout à la fois de favoriser la collecte de l'impôt et de lutter contre les distorsions de concurrence. Afin que les plateformes aient néanmoins le temps de s'adapter à cette nouvelle législation, le Gouvernement avait présenté un sous-amendement, qui avait été adopté par l'Assemblée nationale, visant l'entrée en application du dispositif au 1 janvier 2019. On a récemment appris qu'une célèbre plateforme de location émettait des cartes de paiement prépayées pour détourner

la procédure SANDIA. Un bilan de cet audit sera transmis par la Caisse nationale d'assurance vieillesse à la Direction de la sécurité sociale. Dès lors que la Direction de la sécurité sociale disposera de ces chiffres, le Gouvernement pourra les transmettre au Parlement.

La taxe spéciale additionnelle, la TSA, est un instrument de redistribution des ressources entre les professionnels du cinéma, destiné à favoriser la modernisation des salles et à soutenir la production de films français en passant par une mutualisation des fonds. Mise en application aux Antilles, en Guyane et à La Réunion depuis le 1 janvier 2016 avec une progressivité sur six ans, la TSA constitue une menace sérieuse pour la pérennité de la filière cinéma dans ces territoires si son taux- 10,72 % à terme -n'est pas adapté aux réalités locales. Cet amendement vise donc à instaurer un taux réduit et progressif de TSA à 4,29 % jusqu'en 2022 pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion et à maintenir le taux de 3 % pour la Guyane.

n'est pas intégrée dans l'amendement d'équilibre que je vous présenterai. Je prends bien sûr l'engagement que toutes les conséquences seront tirées lors de l'examen du texte en seconde lecture. L'examen de la seconde partie du texte vous a conduits à rejeter les crédits de cinq missions du budget général, au rang desquelles figurent la sécurité, la justice ou l'agriculture, ce que je regrette. En effet, nous savons tous qu'il n'est pas réaliste de procéder de la sorte pour faire des économies. Je sais pertinemment que personne parmi vous n'entend cesser de rémunérer les policiers et les gendarmes. Cela me permet de vous rappeler que le Gouvernement a précisément fait le choix d'ajuster ces dépenses au moyen de réformes structurelles et documentées plutôt que de procéder par rabot. En outre, le Sénat a amputé de 300 millions d'euros les crédits consacrés à l'aide médicale de l'État ou a encore augmenté de manière forfaitaire le temps de travail dans la fonction publique : en l'absence de documentation précise, la portée de ces votes demeure faible. Au total, et bien que cela soit peu réaliste, comme je viens de l'indiquer, le déficit budgétaire mis en cohérence avec l'ensemble des votes est révisé à la baisse de 51,4 milliards d'euros par rapport à l'équilibre voté en fin de première partie par votre assemblée. C'est la raison pour laquelle nous déposerons cet amendement d'équilibre. Le Gouvernement

en dégradation de 3,3 milliards d'euros par rapport à l'équilibre budgétaire présenté dans le projet de loi de finances. Pour être tout à fait précis, ces 3,3 milliards d'euros incluent les conséquences du vote sur le premier